Par mes chers collègues, Madame la Ministre à toutes et à tous mes meilleurs voeux pour ce millésime 2022, la séance est donc reprise l'ordre du jour appelle le débat sur la politique mise en place par le gouvernement pour conforter la souveraineté maritime française sur les océans et garantir nos intérêts économiques et stratégiques, c'est une demande du groupe des Républicains, la parole est donc tout d'abord, l'orateur du groupe, qui demande ce débat monsieur Alain Cadec pour 10 minutes chers collègues.

Madame la présidente. Madame la Ministre de la mer. Mes chers collègues. En préambule, je souhaiterais remercier mon groupe pour l'inscription de ce débat à l'ordre du jour car les enjeux qu'il recouvre sont essentiels pour l'avenir de la France. Ces enjeux sont globalement bien connu et bien compris de toutes les parties prenantes et de tous les acteurs politiques. Il concerne le maintien de notre souveraineté territoriale et de nos droits exclusifs dans les zones concernées ainsi que notre capacité à assurer une surveillance appropriée de ces espaces. Cela a pour but d'empêcher les violations et les activités illicites et à nous mettre en mesure d'exploiter durablement toutes leurs potentialités économiques. Qu'il s'agisse de l'exploitation des ressources halieutiques et énergétiques et minérales ou des multiples autres activités qui ont pour cadre le milieu marin. Les défis considérables qui correspondent à ces enjeux sont de nature éminemment géopolitique. Et concerne tout simplement la place et le rôle de la France dans le monde. Celle qu'elle occupe actuellement, bien sûr, et celle qu'elle Aspire à occuper dans les décennies qui viennent. Ils exigent pour y faire face, une véritable vision stratégique à moyen et long terme. Et une approche nécessairement holistique des problématiques très variées que recouvre une politique maritime digne de ce nom. C'est tout le sens, Madame la Ministre de votre ministère, ce ministère de la mer qui est en charge de cette belle mission sans pour autant maîtriser directement tous les aspects et tous les leviers. D'ailleurs, ceci n'est pas une critique personnelle, bien entendu, tous les gouvernements successifs ont été confrontés à la même difficulté s'agissant de la politique maritime de notre pays. Comment assurer la cohérence de l'action publique en la matière, compte tenu de la grande diversité des décideurs politiques, des niveaux d'intervention des administrations et des parties prenantes concernées. Et comment obtenir la mobilisation de moyens financiers, humains, logistiques suffisants au service de cette politique, compte tenu de l'énormité des besoins. Un cadre qui n'est sans doute pas parfait mais qui a le mérite d'exister, a été défini en février 2017 sous la forme d'une stratégie nationale pour la mer et de littoral autour de 4 grands objectifs. Le développement de l'économie bleue durable le bon état écologique du milieu marin. La préservation d'un lecteur d'un littoral attractif. Et enfin, le rayonnement de la France. Un quinquennat s'étant écoulé depuis l'adoption de cette stratégie, où en est-on aujourd'hui dans sa mise en oeuvre effective des succès remportés des difficultés rencontrées ou des nouveaux défis identifiés. Pour ma part je voudrais saisir l'occasion de cette intervention pour signaler 2 grands sujets d'inquiétude. Le 1er porte sur le maintien, voire la défense de notre souveraineté et de nos droits exclusifs sur les espaces qui constituent le domaine maritime de la France. Le défi est évidemment très grand compte tenu de l'immensité de ces espaces. Près de 11 millions de kilomètres carrés au total, c'est le 2ème domaine maritime mondial, je ne vous apprends rien dont 97 % sont liés à nos départements et collectivités d'Outre-Mer. Ainsi qu'aux Terres australes et antarctiques françaises, or le contexte géopolitique dans certaines des régions concernées est devenue particulièrement tendue. Notamment le bassin indo-Pacifique où la Chine a crû de manière spectaculaire, ses capacités militaires et hésitent de moins en moins, a affirmé ses prétentions hégémoniques. Comme le souligne le rapport de nos collègues Pascal Alizart et Gisèle Jourda. Que le dernier référendum sur l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, prévu depuis 98 se soit tenu alors que planent de telles menaces de la part de la Chine et que la France vient de se voir exclues spectaculairement. De l'alliance constituée par les États-Unis avec l'Australie et le Royaume-Uni est certes une coïncidence malheureuse. la façon dont ces dossiers ont été gérés par le gouvernement et la manière dont il a communiqué sur ces sujets n'ont pas envoyé, selon moi, les bons messages à nos partenaires et concurrents. Concernant la détermination de la France à rester un acteur majeur dans l'indo-Pacifique au contraire. Le sentiment qui prévaut est que la France a été sur le dossier du référendum pour le moins passive voire absente et sur le dossier des sous-marins que ces fait simplement rouler dans la farine. De manière plus générale, se pose la question de la capacité pour notre Marine nationale d'assumer une surveillance efficace de toutes les composantes de notre domaine maritime pour décourager ou répondre à toute tentative d'intimidation militaire ou de prises de position territoriale mais aussi pour lutter contre la piraterie. Notamment dans l'océan Indien et pour détecter et sanctionner toutes les activités illicites, notamment en matière de pêche illégale. Notre Marine nationale un légitime, objet de fierté. Pour les Français d'ailleurs de même d'ailleurs que notre administration maritime. Pouvez-vous nous assurer, Madame le Ministre, cependant que les moyens dont elle dispose sont suffisants pour accomplir toutes ses missions et se développer comme il se doit dans les années à venir. La question de l'intégrité de notre domaine maritime comporte aussi des aspects juridiques et diplomatiques. Pour empêcher des revendications intempestives de la part de pays riverains, la France doit poursuivre ses efforts de délimitation territoriale dans toutes les zones où c'est cette délimitation n'est pas encore fermement établi, elle doit aussi éviter. De donner à certains de ces pays à travers des accords internationaux un accès trop généreux des hauts sur lesquels ceux-ci pourraient être tenté ensuite de revendiquer des droits. Je salue au passage la vigilance et l'action de notre collègue Philippe Folliot concernant l'atoll de Clipperton est de l'île de Tromelin. Pour alerter sur une certaine négligence de la France dans la protection de ses intérêts. Mon 2ème sujet d'inquiétude porte sur la capacité de la France d'exploiter au mieux toutes les ressources et opportunités économiques offertes par son domaine maritime. Comme vous le savez, mon mandat précédant au Parlement européen, m'a amené à me consacrer, particulièrement à la politique de la pêche. Et dans ce seul secteur, bien des choses pourrait être dite au sujet par exemple de l'évolution de la PCP vers toujours plus de contraintes et de restrictions pour nos pêcheurs sans se préoccuper des conditions dans lesquelles sont pêchés les millions de tonnes de produits de la mer importés chaque année dans l'Union européenne. Petit aparté. S'agissant des retombées très négatives du Brexit sur la pêche française, le gouvernement a ne semble-t-il manqué de fermeté face à la passivité de la Commission européenne. Dans le rôle de fait dont le rôle est de faire appliquer l'accord. Et non de céder aux injonctions des Britanniques. Mais la problématique est évidemment plus large et s'étend également aux ressources énergétiques et en matières premières. Sans compter tous les secteurs de service et les industries navales, le tout représentant un ensemble d'activités économiques liées à la mer très important à la fois en termes de PIB et en termes d'emploi. Beaucoup des activités en question nécessite d'être soutenu et développé, c'est notamment le cas pour ce qui concerne les ressources minérales présente dans les fonds marins et sulfure nodules poly-métalliques, les encres hautement cobalt Qui représente un immense potentiel dans un contexte global de raréfaction et de renchérissement des matières premières mais dont la plupart des gisements doivent encore être localisés et sont d'accès difficile. Une course est déjà bien engagée entre les grandes puissances maritimes pour l'accaparement de ces ressources, il importe madame le Ministre que la France ne prenne pas de retard en la matière. Cet exemple doit aussi nous rappeler l'importance de la science et de la recherche fondamentale et appliquée pour une meilleure connaissance des fonds et du milieu marin. L'occasion de saluer l'action d'Ifremer, qui incarne l'excellence française en la matière, mais dont les projets doivent s'inscrire dans une véritable vision stratégique. Disposer de financements ça suffisant et autant que faire se peut, le secteur privé. Je voudrais conclure sur cette question des ressources et opportunités économiques offertes à la France par son vaste domaine maritime en mettant en garde contre certains excès liés à la préoccupation écologique. Je relève que des 4 grands objectifs de la stratégie nationale pour la mer et le littoral définie en 2017, comme je le disais tout de suite 3 sont entièrement ou en grande partie lié à la protection de l'environnement. Alors, ces objectifs sont évidemment légitime mais leur poursuite ne doit pas occulter selon moi la nécessité pour la France de donner la priorité à la poursuite de ses intérêts stratégiques et économiques dans un contexte global ou d'autres grandes puissances maritimes ne s'embarrasse pas toujours des mêmes contraintes. Je pourrais pas me dire le contraire, Madame la Ministre, dans plusieurs rapports sur la pêche, aussi bien au Parlement européen que dans cette assemblée, j'ai utilisé en paraphrasant Staline. L'expression de durabilité dans un seul pays. Pour souligner la faiblesse intrinsèque de politiques qui font reposer sur la France ou sur la seule Union européenne, le poids des efforts à consentir pour assurer la protection du milieu et la préservation des ressources. La France dans la définition et la mise en alerte de sa stratégie maritime ne doit pas tomber dans ce travers, il importe donc que son action résolue en faveur du milieu marin s'exerce avant tout dans le cadre des organisations internationales multilatérales et régionales compétentes en s'assurant en permanence d'un effort partagé, partagé équitablement par tous les pays concernés, plutôt que de manière unilatérale. Alors, à quelques mois d'un nouveau quinquennat chers collègues, il ne il était en tout cas, opportun pour cette assemblée de faire le point en prenant un peu d'altitude et de recul sur ses importantes thématiques afin d'assurer, pour utiliser une métaphore maritime que le cap est le bon et que la barre est fermement tenue. Merci mon cher collègue. Dans la suite des débats, la parole est au groupe et nous commençons par Joël Guerriau, qui représente le groupe des indépendants, vous avez 5 minutes chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Le pays entretient un lien particulier avec la mer, notre histoire, nous a conduit à parcourir, a traversé tous les océans, ainsi le territoire national de la République française se trouve aussi bien en Amérique du Nord, dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, dans les océans Indien et Pacifique mais aussi en Antarctique, cette diversité est une chance pour notre pays, nous nous réjouissons à cet égard que les néo-. Calédonien est fait pour la 3ème fois le choix de rester français en décembre dernier. La délégation territoire sénatoriale aux outre-mer a produit un grand nombre de rapports extrêmement riche en matière de préconisation, je me souviens, pour ma part, de l'un d'entre eux, dont j'avais été le coauteur en 2014 et dans lequel nous préconisions d'instituer un ministère de la mer aussi, je me réjouis de votre présence, Madame la Ministre, nous avions plusieurs recommandations concernant la promotion aux échelons national, européen et mondial. D'un cadre normatif pour une économie bleue durable, notamment par la prise en compte de la fragilité du milieu marin dans le code minier. Quelles sont les avancées sur le plan international, Madame le Ministre, où en est la convention de Montego Bay. La Chine qui a ratifié le texte, on piétine les principes et les États-Unis, qui ne sont pas signataires eux défendent les mêmes principes, nous préconisons aussi la restructuration de nos activités marines en filière intégrée de la recherche jusqu'aux activités marchandes, avons-nous. Progresser à ce sujet le domaine maritime revêt pour la France une importance toute particulière au vu de sa présence sur l'ensemble du globe, ce domaine est une richesse que beaucoup nous envient et que nous devons savoir mettre en valeur. Pour cela, il est essentiel de connaître avec précision la composition de ces espaces, le Service hydrographique et océanographique de la marine, le CHUM et l'un des principaux piliers de cette connaissance. Le développement d'un prototype d'un robot sous-marin devrait nous permettent. De nous doter d'une capacité d'investigation à grande profondeur, à la fin de cette année, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, les Frommer a mené plusieurs études visant à améliorer la connaissance de nos fonds marins mais force de constater qu'il nous reste encore beaucoup à découvrir, nous avons eu l'occasion de le regretter, nous l'avons dit le retard qui a été pris par le programme, capacité de. Océanographique du futur à l'heure où le monde, les yeux rivés ont les yeux rivés sur la zone Asie-Pacifique, les Russes et les Chinois se montre très actif en la matière est prête une grande attention à ce milieu qui voit passer l'essentiel du commerce mondial, ainsi que d'importants câbles de télécommunications, il est temps essentiel que notre pays ne prenne pas de retard en la matière au-delà de la connaissance, il est également primordial que la France dispose de la maîtrise de ses eaux, nous avons vu certains pays tentés de nous déstabiliser, là où nous avons des territoires d'Outre-Mer nous envoyons d'autres tester régulièrement notre vigilance au large de nos côtes, la France dispose d'une marine de 1er ordre, le gouvernement a maintenu les efforts prévus par la LPM et nous nous en félicitons, notre pays est l'un des rares puissance mondiale disposant d'une dissuasion nucléaire sous-marine silencieuse et intellectuelle, un des télés tables nous voyons s'accroître les menaces, la stratégie de durcissement de préparation à la haute intensité répond bien à cette réalité, le budget de la défense doit être à la hauteur des missions qui sont confiées à nos armées, ces efforts doivent nous assurer la supériorité, notamment dans le domaine maritime, les sous-marins SNA de classe Barracuda figurent parmi les meilleurs de leur catégorie. Combiné aux autres moyens de la marine, ces bâtiments nous permettent d'assurer des missions de surveillance ainsi que de protéger la France de ses intérêts partout dans le monde la regrettable décision de l'Australie. Revenant sur sa commande de sous-marins français pour finalement naviguer sur des bâtiments américains n'enlève rien à l'application de notre pays dans cette zone, nos territoires ultramarins et notre coopération avec les acteurs de l'espace indo-pacifique, nous y inscrire dans la durée. J'ai eu la chance récemment de visiteurs n'pas une sorte satellitaire de l'Union européenne, j'ai pu voir des grappes de bateaux de pêche chinois, est ce que. C'est par des frégates pour ratisser les fonds de l'indo-Pacifique cette réalité doit nous inciter à renforcer notre présence dans cet espace nous astreindre à l'exemplarité en matière environnementale, la France participera à l'histoire de cette région qui compte parmi les plus stratégiques de la planète. La Chine a compris que pour dominer le monde, il faut être une grande puissance maritime. Le général De Gaulle en 1969 n'affirma-t-il pas que les États chercheront à dominer la mer pour en contrôler les ressources, nous y sommes, il est de notre responsabilité, madame la Ministre de préserver nos intérêts en se donnant tous les moyens pour le faire, merci de votre attention. vous avez 5 minutes chers collègues. en 1994 Jacques Chirac disait : les Français aiment la mer, mais ils la connaissent mal ces mots reste d'actualité, près de 30 ans plus tard, même si la France possède le 2ème domaine maritime mondial après les États-Unis, les gouvernements successifs ne semblent pas avoir pris la mesure de ce bien stratégique pour notre économie et notre souveraineté et cela malgré le récent Fontenoy du maritime, la crise du coronavirus les dérèglements climatiques et le Brexit ont accentué la fragilité de l'économie maritime française et donc de sa souveraineté, car il n'y a pas de souveraineté maritime sans une véritable ambition pour notre marine française et donc une ambition aussi portuaire et c'est sur ce sujet que je voudrais intervenir ce soir en effet, l'année dernière, le Sénat et qui est porteur d'une recommandation sur la stratégie nationale portuaire, nous pouvons nous féliciter collectivement que ce rapport est plus inspiré de gouvernement comme l'expliquer monsieur le 1er ministre au dernier comité interministériel de la mer ou en janvier 2021, mais à l'aube de la fin de ce quinquennat l'urgence est de mise, il faut aller plus loin et s'inspirer directement des travaux de l'Institut Montaigne qui décide une véritable ambition pour la stratégie maritime française au-delà des 1,5 milliard d'euros pour les ports de l'axe Seine des 650 millions d'euros attribués au volet maritime dans le plan de relance et de la fusion des ports, notamment de l'axe Seine les faiblesses de nos grands ports maritimes qui sont la base de notre stratégie maritime, et notamment des grands ports métropolitains et ultramarins sont bien identifiés, porte de l'Europe, passage incontournable nos ports font face à un défi de fiabilité et d'efficacité, la première raison est connue, c'est le climat social qui, depuis 2016 est assez instable, notamment avec plusieurs opérations porcs morts ces actes condamne peu à peu chaque jour, nos ports face à la concurrence de nos voisins, notamment de de l'hinterland du nord de l'Europe, de plus, notre internaute national est bien trop mal reliés et malgré l'E-Mode théâtre, à proximité de l'Île-de-France, trop de route, pas assez de trains et de transports fluviaux, la mer est ce qui nous relie au monde entier, mais sa frontière la terre doit être le bras armé efficace notre politique de souveraineté maritime et non son handicap, c'est la condition de notre survie au moment où le Brexit impacte nos pêcheurs, nos ports et nos échanges internationaux, vous le comprendrez, il faut aussi un plan Marshall du maritime en France pour avoir une véritable ambition relatives à notre souveraineté nationale, c'est ce que le Sénat appelle de ses voeux, en effet, malgré une véritable stratégie d'aménagement du territoire vers le et le report modal vers le ferroviaire et le fluvial, il est important de développer aussi ces modes de reports notamment d'un point de vue économique mais aussi écologique, taxe doit être prioritaire au moment où se crée notamment des axes comme le canal Seine Nord qui reliera les ports du nord de l'Europe à l'internaute. Le rapport du Sénat sur réarmer nos ports préconisé un triplement des aides me combiné au port aux transports, et ce malgré une augmentation prévue dans le plan de relance, nous sommes loin du compte pour les ports français qui sont essentiels au développement de notre stratégie n'maritime française, enfin, dans le cas d'un Brexit dur et mon collègue à la Cadac Cadec que la signaler des des relations que nous entretenons avec les Britanniques, il est urgent aussi d'expérimenter le concept de port franc afin de rivaliser avec les ports anglais, c'est cette nouvelle bataille que nous devons gagner pour pour maintenir cette hégémonie française et notre souveraineté sur l'ensemble du notre stratégie maritime en lien avec les collectivités locales, les zones franches porteurs peuvent être un levier pour maintenir nos ports à flot ces idées et ces dispositifs existaient déjà, ils sont possibles, déjà annoncé l'air lors des 2 derniers 6 mais aussi aujourd'hui non suivies d'effet, il est temps, Madame la Ministre qu'elles aboutissent dans les meilleurs délais, face à la affaire férocité pardon croissante de la compétition internationale dans ce secteur, le renforcement de l'attractivité de nos ports et plus que jamais un impératif pour doter la France des moyens d'agir efficacement pour que la souveraineté maritime française soit maintenue sur nos océans, je vous remercie. Merci, cher collègue à la parole est à présent à notre collègue Jacques Fernique du groupe écologiste pour 5 minutes. merci madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Les changements que nous avons déjà provoqué dans le système océanique perdureront pendant des siècles et aggrave la crise climatique, ce sont les mots de Dan de l'Union internationale pour la conservation de la nature, la prise en compte de l'océan est effectivement essentiel si l'on veut parvenir à atteindre, à la fois les objectifs climatiques de l'accord de Paris et les objectifs pour la biodiversité. La France, on l'a dit qu'il possède le 2ème espace maritime au monde, un rôle déterminant à jouer pour la transition écologique du monde maritime notre groupe ça n'étonnera pas, ne partage pas là-dessus, l'opinion de notre collègue Alain Cadec sur ce qu'il considère, pour reprendre ses mots comme des excès liés à la protection écologique ces enjeux de durabilité sont d'autant plus important, a relevé que la réalité économique du monde maritime pèse fortement le secteur maritime français représente davantage d'emplois que l'industrie automobile. Nous interrogeons par notre débat de ce soir, notre politique nationale pour conforter leur souveraineté maritime et garantir nos intérêts économiques et stratégiques, nous savons tous cependant combien la politique à mener ne peut être une logique strictement national combien les capacités européennes et la coopération internationale sont déterminantes en la matière, l'océan est aussi le jeu des puissances qui se disputent les espaces maritimes depuis l'Antiquité, la zone indo-Pacifique est ainsi fortement marquée aujourd'hui par l'affirmation de la Chine, notre indépendance numérique aussi se joue au fond des océans d'autres pays qui étaient en pointe sur la télécommunication sous- marine a besoin aujourd'hui d'une dynamique européenne forte, si nous voulons contrer aujourd'hui la domination des Gafam. Au total, le défi de la France et de tenir son rang et ses responsabilités, particulièrement pour la mise en oeuvre et de cette transition écologique par sa présence dans les océans par ses territoires d'Outre- mer par de solides Liens de coopération internationale et ainsi contrer l'effondrement de la biodiversité, d'abord par la lutte contre la surpêche particulièrement la pêche illégale pour laquelle le bras de fer avec la Chine doit être ferme comment assurer cette transition écologique, alors que les tensions géopolitiques s'amplifie que les enjeux géo-économiques et stratégiques sont multiples, que les intérêts d'exploitation économique à courte vue, sont si puissants, n'est-ce national d'exploration et d'exploitation des ressources minérales dans les grands fonds marins présenté par le secrétariat général de la mer il y a un an et confirmé dans le plan d'investissement France 2030, a annoncé la couleur : le moins que l'on puisse dire, c'est que ces orientations ont fait tâche au lendemain du congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature, le président de la République a dit clairement son opposition avec la proposition de moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins portés par l'UICN dévalorisant ainsi d'une certaine façon, ses propres déclarations en faveur de la protection des océans nous regrettons pour notre part que le gouvernement n'exclut pas la possibilité d'exploiter des ressources minérales dans les zones protégées une telle gestion ne pourrait être rondement qualifiée de durable, entendons les préoccupations exprimées par les scientifiques pour qui la perte de la biodiversité sera inévitable si l'activité minière des grands fonds marins est autorisée, les avantages à long terme d'un océan dépassant de dépasse de loin les opportunités à court terme, offertes par l'exploitation minière des fonds marins, la demande de minerai nécessitera de plus en plus des processus efficaces d'économie circulaire encourageons avant tout, l'innovation, le recyclage et la réparation plutôt que de miser sur le mirage de l'économie bleue engager résolument notre stratégie maritime dans la transition écologique, loin de freiner la France est gage d'opportunités économiques sociales géopolitique par quels engagements y parvenir : d'abord en crédibilisant l'objectif de neutralité carbone du transport maritime à l'horizon 2050 c'est ce qu'ont déjà initié nos voisins scandinaves ont protégeant ensuite effectivement au moins 30 % de l'océan, au moyen d'aires maritimes protégées, les résultats des réserves marines quand elles sont sérieuses et strict sont spectaculaires, déjà même à court terme, à condition de n'effectuer aucun prélèvement de plénitude des espèces peuvent être rapidement retrouver des réserves marines efficace, c'est bien sûr la reconquête de la biodiversité, c'est bien sûr aussi le repeuplement des zones de pêche l'océanographe François Sarano nous l'a dit clairement devant notre commission développement durable, il est nécessaire de transformer les pêcheurs exploitant empêcheur gestionnaire, passer d'une logique de subventions à la destruction, à une logique de rémunération à la gestion collective le chalutage profond doit être bannie c'est aujourd'hui encore loin d'être le cas, donc en 5 minutes, je voulais insister sur cet enjeu majeur, plutôt que de passer en revue tous les volets du débat qui nous ont proposé, je laisserai le monde ma conclusion à Dan l'affoler, à nouveau, la protection de l'océan est affaire de survie humaine, il s'agit d'en prendre acte. Merci, cher collègue, la parole est à présent au président Laurent du groupe communiste. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, avec 11 millions de kilomètres l'espace maritime français représente le 2ème territoire maritime le plus important du monde, que faisons-nous de cette immense responsabilité aux enjeux multidimensionnel, pas seulement au vu de la fenêtre étroite qu'énonce le débat demandé ce soir par le groupe Les Républicains, je cite : garantir nos intérêts économiques et stratégiques mais vu avec la hauteur qui sied au rôle que devrait jouer la France pour la protection de ce bien commun mondial stratégique pour l'avenir de la planète, n'oublions pas les mots du poète, la Terre est bleue comme une orange, bleue comme la masse des océans il y a bien 2 manières d'entrer dans ce débat, la recherche de la puissance stratégique, économique, militaire qui place inévitablement mers et océans, au coeur de la compétition mondiale, ou alors la prise de conscience du rôle nouveau que peuvent jouer mers et océans dans la construction d'un futur durable pour l'humanité toute entière, je crois que la France sans naïveté aucune sur les rivalités de puissance qui se joue sur les maires devraient choisir la seconde approche, elle nous donnerait plus d'ambition pour faire de notre souveraineté maritime : un atout au service du bien commun mondial, elle nous ouvrirait des champs immenses d'alliance et de coopération nouvelle l'approche dominante de la mer et des océans, reste aujourd'hui calqué sur la conception de la mondialisation et des échanges historiquement construite autour du contrôle politique, économique et militaire des grandes routes maritimes géostratégique reliant de port en port les zones de ressources et de matières premières aux riches nations occidentales nous prétendons maintenir à tout prix ce contrôle alors que des régions entières nouvelle demande à contrôler leurs ressources et à disposer elle aussi d'un droit d'accès à ces grandes voies de circulation mondiale et d'autre part, réchauffement climatique et bouleversements géopolitiques redessine la carte du monde et font surgir de nouveaux enjeux résultat notre vision de la sécurisation de l'espace maritime est doublement dépassée, elle est auto-centré sur une vision dépassée de nos intérêts et elles sous-estiment les nouvelles ambition nécessaire pour une stratégie maritime au service de la sécurité globale, planétaire, tout le monde, par exemple la place grandissante des enjeux de protection civile et de protection de l'environnement dans la mission même de nos moyens militaires maritimes, il y a beaucoup d'exemple en la matière, tout montre aussi que, dans ce cas comme dans bien d'autres, la faillite de la gestion européenne ou mondiale de ces crises et présente, rappelons-nous, par exemple pour le secours aux migrants en mer le sabordage de l'opération Sophia que nous avions tenté de construire et séquences jusqu'à aujourd'hui, qui font des routes de l'exil, les routes migratoires les plus dangereuses du monde, selon les ONG en mer, notre priorité, pourtant, on n'est semble-t-il pas là notre approche sécuritaire reste avant tout militaire mais là aussi, pour quel résultat on Europe par exemple, renouveler le renouvellement des moyens de patrouilles militaires bute sur le choix allemand acheter plutôt Boeing que Dassault tournant une fois encore le dos à l'autonomie au européenne et dans l'indo-Pacifique : États-Unis, Royaume-Uni nous ont écarté sans ménagement du contrat des sous-marins australiens, faut-il dès lors, courir après l'escalade à la confrontation militaire, je crois que ce serait une folie, c'est une autre conception qu'il convient d'déployés. Mon camarade et collègue Jean-Paul Lecoq à l'Assemblée nationale, soulignait l'ampleur des actions stratégiques à conduire pour protéger et développer notre espace maritime la surveillance le sauvetage, la lutte contre la piraterie le brigandage maritime contre les pollutions de toutes sortes, cuir criminelle, accidentelle pour la dépollution des océans pour la protection des ressources halieutiques pour l'est donc à de catastrophe naturelle. Nous devons tenir notre rang au service de la sécurité globale et les domaines où il convient d'investir sont nombreux et ils sont à notre portée, si nous mobilisons nos atouts nationaux et des multiplions les coopérations internationales pour le lutter contre les grands défis écologiques, les grandes invasions biologiques Maryline, par exemple, pour développer une nouvelle conception de la pêche, axée sur la protection des ressources halieutiques pour le réinvestissement dans la construction navale incroyablement délaissée dans notre pays, alors que nous sommes le 2ème espace maritime mondial pour le retour d'un État stratège pour le développement de nos ports en métropole comme en outre-mer pour le développement des énergies marines renouvelables c'est au service de la protection de cette nouvelle conception de notre politique maritime que nous devrions réfléchir. Un dernier mot sur une question qui vient d'être évoqué les fonds marins regorge de minerais précieux de métaux rares, de nombreux États se font la course pour s'accaparer ces ressources stratégiques lors du dernier congrès de lui CM l'Union internationale pour la conversation conservation 100 des États et 95 % des ONG ont voté en faveur du moratoire sur l'exploitation de l'exploration minière des fonds marins, la France s'est abstenu, nous proposons au contraire que la France propose de reprendre cette proposition pour ce moratoire et pour signer ensemble un traité international visant à protéger les fonds marins de toute exploitation. je vous remercie. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les conflits en indo-Pacifique les tensions en Arctique en mer Noire, ou en mer de Chine des problématiques d'exploration marine ou encore la rivalité franco-britannique sur les accords de pêche post-Brexit sont autant de sujets qui illustrent l'importance mais aussi l'aspect multi-dimensionnel des enjeux maritimes du 21ième siècles depuis la Grèce antique, les nations les plus puissantes sont maritime. Comme cela a déjà été rappelé la France détient le 2ème plus vaste espace maritime du monde avec plus de 10 millions de kilomètres carrés que nous devons en grande partie à nos outre-mer. La sûreté de cet espace stratégique reste essentiel pour notre souveraineté et notre Marine nationale déployé sur tous les océans à cet effet. Une partie non négligeable de notre économie, de notre industrie et de notre diplomatie est tournée vers la mer dans la vive compétition mondiale dont les ressources océaniques et la sécurisation des intérêts nationaux sont aujourd'hui l'enjeu : la France dispose d'atouts pour asseoir et développer sa vocation maritime. à ce triplé notre stratégie nationale de sûreté des espaces maritimes articulé avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral, entrée en vigueur en 2017 doit constituer un socle solide de réflexion pour que la France relève les défis qui garantiront à la fois l'essor et la survie de notre puissance maritime. Compte tenu de l'étendue du sujet, je ne développerai que certains points qui me semble essentiel. Tout d'abord la défense de nos intérêts stratégiques entre tension et convoitise : les défis de souveraineté, nous espace maritime ne manquent pas plusieurs contestations portent sur les délimitations de notre espace et oppose des États tiers à la France. La remise en cause de l'extension de certaines aides les manoeuvres ou de bâtiments militaires étrangers, le développement d'activités illicites dans nos eaux doivent nous obliger à une certaine fermeté pour faire valoir nos droits et assurer une surveillance de ces zones. Autre sujet crucial pour nos intérêts stratégiques, celui des routes maritimes aujourd'hui plus de 70 % de nos importations et de nos exportations, ainsi que le ravitaillement de nos territoires d'Outre-Mer et de nos forces militaires empruntent des voies maritimes, l'accessibilité des grands axes et donc stratégique et vital à court terme, ces derniers ne devrait pas être bouleversé cependant à moyen terme, compte tenu de la baisse des besoins en pétrole brut au profit des produits raffinés et l'augmentation des besoins en gaz naturel l'importance stratégique de certaines routes pourraient évoluer, il me semble important aujourd'hui de mettent l'accent, avec les acteurs privés sur l'analyse des évolutions des flux stratégique et d'adapter notre stratégie à toute nouvelle menace sur les routes existantes ou futures. Enfin ce sujet des routes maritimes, il convient de souligner la décision de la CMA CGM, qui s'interdit d'emprunter les routes du Nord pour favoriser la protection des écosystèmes fragiles de l'Arctique, nous ne pouvons que saluer Madame le Ministre, cette décision, respectueuse de l'environnement, à ce titre, la France est-elle exprimée pour inviter les armateurs étrangers agir également dans ce sens. 2ème point que je souhaitais évoquer nos intérêts économiques, certes, la France occupe une place centrale dans de nombreux secteurs de l'économie maritime. Je pense par exemple à la construction avec les chantiers aux transports avec des armateurs présents dans les différents secteurs ou encore aux entrepreneurs dans les services de travaux maritimes qui se développe avec l'économie bleue. La marine marchande, est aujourd'hui un instrument de souveraineté pour garantir nos approvisionnements et nous nos exportations très dépendant du transport maritime. Pourtant depuis bien trop longtemps ce secteur manque d'ambition commune pour garantir nos intérêts. C'est pour cette raison, Madame la Ministre, que je salue le travail mené dans le cas du Fontenoy du maritime visant à à quoi, la croate, pardon la compétitivité du pavillon français pour renforcer la place économique et industrielle maritime française, il demeure cependant un problème central, celui de nos places portuaires qui continuent d'accuser un retard par rapport à nos voisins européens, la puissance économique d'une nation se mesure par la présence ou non de très grands ports de commerce, aucun pays ne peut poursuivre une ambition stratégique, économique et comme je écologique sans cela la modernisation en cours nécessitent encore des investissements d'infrastructures lourds mais aussi une diversification des activités portuaires enfin un mot sur les enjeux liés à la pêche, la crise des licences post-Brexit a une fois encore mis en lumière le poids économique de ce secteur, mais aussi et surtout le fort attachement des Anglais à leur souveraineté maritime. Au-delà des considérations politiques, une réalité s'impose à travers le monde la demande de poisson étant croissante et les ressources halieutiques sauvages de plus en plus rares, l'accès aux différentes zones de pêche et aquacole devient de plus en plus stratégique ainsi l'enjeu concerne la sécurité alimentaire de la population et la nécessité de fournir au marché au marché français, l'apport en protéines issues du milieu marin, nous devons continuer à défendre et nos intérêts, notamment en coopération avec nos collègues européens ceci m'amène au dernier point que je souhaite évoquer l'engagement de notre pays pour la protection de la biodiversité et de la ressource, mais aussi pour le développement d'une activité économique durable essentiel notre souveraineté maritime réside dans notre capacité à protéger nos ressources face au dérèglement climatique à la pollution des océans, la protection des mères est devenue un enjeu majeur pour la France, qui a développé un programme de protection de ces aires marines en France métropolitaine, comme dans les Outre-mer ces aires marines protégées poursuivent un but de préservation de la nature. Cet objectif de protection n'est pas exclusif d'autres objectifs, qui envisage-t-on Madame le ministre à long terme comme projet et pourra venir pour ces zones, plus globalement, les secteurs de la mer en tant, joue un rôle dans la transition écologique de la France vers le développement durable, contribue à une économie prospère et à la préservation de la mer, l'État partage bien évidemment cette vision. La presse se fait actuellement l'écho d'une réorganisation des services de l'État, le gouvernement prévoit de fusionner la direction des affaires maritimes et la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture pensez-vous Madame la Ministre, que cette nouvelle direction de la mer aura les moyens et sera répondent à la préservation de notre souveraineté en alliant les enjeux économiques et environnementaux, l'espace maritime est non seulement une composante constitutionnellement affirmés de la République française, mais il est aussi un vecteur de l'autorité du rayonnement de la France sur la scène mondiale, notre pays est un des rares États au monde, riverain de 3 océans Atlantique, Pacifique et Indien, nous devons redoubler d'effort pour conforter nos souveraineté maritime en protégeant nos ressources pour des raisons politiques, économiques et environnementales, tout en travaillant à garantir la liberté de circulation sur les mères dont on sait combien elle est aujourd'hui menacée. Merci, cher collègue, la parole est à présent André sénateur représentant le groupe RDSE, vous avez 5 minutes chers collègues. Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, le temps du mari libéraux mais chère à Hugo consensus est-il en passe d'être révolue l'idéal de liberté propre l'espace maritime se heurtent de plus en plus à la compétition qui se joue en son sein la revue stratégique de défense et de sécurité nationale de 2017 non, c'est clairement l'espace maritime comme un enjeu traditionnel de rivalités entre les grands États, ce que confirme l'actualisation stratégique 2021 qui rappelle les rapports de forces à l'oeuvre dans les fonds marins notre pays en tant que 2ème puissance maritime a le plus à perdre en termes de souveraineté, si rien n'est fait pour que ce All davantage réguler l'activité à la fois économique et stratégique, tirer des mers et des océans, alors Madame la Ministre, nous sommes face à un thème aussi complexe qu'évolutif qui rappelle forcément une multitude qui appelle forcément une multitude de réponses et c'est tout l'intérêt de notre débat et de nos échanges de ce soir tout d'abord, peut-on envisager une planification de la gestion des Verts à l'échelle internationale, comme les États de l'Union européenne aussi emploie poussés par la directive de 2014 la France y trouvait-t-elle son intérêt compte tenu de sa position privilégiée du à ces territoires d'outre-mer, notamment si quelques critères organisées l'exploitation partager bien entendu de façon durable, un espace de haute valeur marchande et stratégique en tout cas la convention des Nations unies sur le droit de la mer doit évoluer afin que les grandes puissances n'imposent pas leur seule règle des règles pas forces sournoise qui aboutissent à vaincre sans combattre, pour reprendre le slogan de la Chine a minima la question sensible est majeure des câbles sous-marins mériterait d'être mieux appréhender sur le plan du droit international, la captation malveillante des données par ce biais, est un de plus en plus courantes en attendant depuis Blaise Pascal, nous savons que l'humanité n'a pas su faire en sorte que la justice soit toujours la plus forte et qu'elle a dû mettre la force à la disposition de la justice, aussi devons-nous disposer d'une force d'action navale imposante entraîner reconnue et donc respectée, c'est ce que représente actuellement notre force Marine à travers ses navires, ses sous-marins ses avions, ses satellites et, bien sûr, ces femmes et ces hommes entraînés et engagé parmi les réponses visant à consolider notre souveraineté maritime et si le multitude si la multi-capacité et préservé par la loi de programmation militaire, c'est la question du pouvoir disposer en permanence d'un porte-avions opérationnel, fer de lance, notre groupe d'action navale indépendamment des contraintes matérielles de maintenance qui doit charpenté notre réflexion les études du second porte-avions sont lancés, on s'assurera que le bison temporel couvre totalement notre besoin qu'une réflexion sur la date de sa mise en service et sur celle du retrait graduel du service actif du Charles-de-Gaulle s'impose donc, aujourd'hui notre marine est incapacité d'assurer notre souveraineté dans les arbitrages maritime de faire respecter le droit international, d'assurer la protection des zones exclusives économiques et d'effectuer des sauvetages en mer, mais qu'elle viendra-t-il en cas de conflit longue et de haute intensité, la question de la présence et de leurs nombres de leur armement et la performance de nos bâtiments qui patrouillent sur et sous les océans se pose et, bien entendu, avait la capacité de nos la mise en perspective cette réflexion passe forcément par notre place dans l'OTAN, pondéré par la nécessité complémentaire d'une eau monte impuissance du pilier européen de défense, la place de la dissuasion nucléaire dans la seule la la France dispose au sein de l'Union européenne doit, dans ce contexte aussi être mais de mais de façon plus générale la souveraineté d'un pays repose aussi sur sa réputation, sa notoriété et sur le respect qu'incarne une nation, une réputation méritée à qui j'ai gagné par ses agissements, nationaux et internationaux et par la richesse par la richesse qu'il s'agisse de la construction de paquebots, à Saint-Nazaire Saint-Nazaire qui a été évoqué qui bien que naviguant sous pavillon étranger contribue à la grandeur de la France, et là, en tout cas la démonstration de son savoir-faire, qu'il s'agisse aussi de la politique d'aide au développement aux pays partenaires par la construction d'infrastructures par son savoir-faire agricole ou encore par la diffusion de sa langue et de sa culture et de son enseignement, la France se porte dans le monde une réputation humaniste, la patrie des droits de l'homme, comme la Grèce, porte l'origine de la démocratie et les États-Unis, le concept de liberté individuelle, si bien que conforter la souveraineté maritime de la France et ainsi garantir nos intérêts économiques et stratégiques passe aussi par la fidélité de nos idéaux de justice et de générosité qui doivent demeurer associé à notre présence maritime sur nos océans et les océans, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent à Martine Filleul, du groupe socialiste, vous avez 5 minutes chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, si notre pays possède le 2ème domaine maritime mondial, plusieurs facteurs fragilisent le plein exercice de la souveraineté française sur ces espaces, d'une part et d'autre part, nos politiques ne sont pas à la hauteur, on ne prenant pas suffisamment en compte cet atout la mer est un espace de rigueur et de liberté, disait Victor Hugo, la réalité est aujourd'hui tout autre plaque tournante stratégique des échanges commerciaux ces étendues deviennent le théâtre de nouveaux affrontements l'exemple récent du refus du Royaume-Uni d'octroyer des licences aux pêcheurs français nous la montrer à nos dépens dans ce dossier, la faible implication de la Commission européenne et l'absence d'appui suffisant de pays amis, a révélé la perte d'influence française au sein de l'Union qui mettent à mal notre souveraineté, nous attendons donc de la présidence française du Conseil Conseil permettent de résoudre cette question de remobiliser nos alliés et de mieux articuler compétences et intérêts nationaux et européens. Le changement climatique ne fera qu'accroître ces tensions politiques en particulier s'agissant de la liberté de navigation et de l'accès aux ressources maritimes en effet l'élévation du niveau de l'eau sous l'effet de la fonte des glaces va impacter significativement la délimitation des différentes zones maritimes et donc l'étendue de la souveraineté d'un État côtier comme le nôtre, nous plaidons donc pour que la France oeuvre non seulement pour limiter le réchauffement climatique mais aussi pour porter ses futurs problématique sur la scène internationale, afin de prévoir les mécanismes de prévention de ces conflits. Au-delà de la géographie notre souveraineté maritime nécessite des infrastructures compétitives sûr et sécurisé au 1er rang desquels figurent les ports, il constitue un outil indispensable pour l'approvisionnement en toutes circonstances de nos Thierry toi la crise sanitaire l'a démontré à l'export, ils permettent la promotion de nos filières d'excellence autour de cet enjeu stratégique, je dirais presque régaliens d'importants défis sont à relever, car malgré plusieurs réformes nos places portuaires accuse un important retard, notamment en raison de faibles investissements si nous saluons les moyens dégagés dans le plan de relance et ceux annoncés dans le 6 maires, ils ne seront pas seuls suffisant pour revenir dans la course. Mais plus que jamais l'économie doit se conjuguer avec les impératifs écologiques pour préserver nos ressources océaniques garantir notre souveraineté maritime, c'est garantir notre accès au plein potentiel des océans qui offre des solutions infini pour l'alimentation, la production d'énergie renouvelable, la technologie et la médecine, or leur richesse sont menacées par l'exploitation du trafic maritime, la surexploitation des ressources, la pollution et le changement climatique, les bénéfices des océans sont par conséquent conditionnée par leur protection et la préservation de la biodiversité, en somme, si l'accès à la mer constitue une formidable opportunité, il implique également une forte responsabilité en la matière, il y a loin de la coupe aux lèvres l'ensemble désert sous protection forte représentent moins de 3 % aujourd'hui si la France s'est fixé un objectif de 10 % en 2022, ce dernier manque de précision dans sa définition par le gouvernement, mais il est aussi largement insuffisant des scientifiques estimant qu'il devait être porté à près de 40 de la même manière, dans le cadre de l'autorisation de l'exploration des grands fonds marins par le gouvernement dans son plan d'investissement 2030, nous demandons à ce que des limites claires soient fixées rapidement pour éviter que l'exploration ne débouche sur des exploitations dommageable les océans sont autant indispensable au développement économique au maintien de la vie sur Terre et à la régulation du climat si concilier ces enjeux contradictoires s'avère de plus en plus difficile, c'est néanmoins le défi que nous devons relever pour garantir notre souveraineté, je vous remercie. Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants, vous avez 5 minutes 6 minutes par nos chers collègues, on sort Nadal. Madame la présidente, madame la Ministre, mes chers collègues, la globalisation et la maritime isolation des échanges dans le monde sont en constante hausse en augmentation, elles sont au coeur des enjeux diplomatiques internationaux nos contemporains, la présidence française du Conseil de l'Union européenne sera l'occasion de mettre au centre des discussions la question de la stratégie de l'Union sur ce point, la France et la 2ème zone économique exclusive au monde, nous sommes le seul pays européen à disposer d'une telle ouverture et nous occupons une place importante dans plusieurs secteurs de l'économie maritime, la construction, le transport, la recherche ou encore l'armement mais malgré cette situation exceptionnelle, l'économie bleue ne représentent que 2 % de notre PIB nos propres potentiel économique maritime a été ces dernières décennies, sous-exploité nos faiblesses sont connus des ports métropolitains peu compétitifs des ports d'outre-mer à l'écart des routes maritimes, fort de ce constat, vous avez agi, Madame la Ministre, dès 2017 vous avez défini un cadre de stratégie nationale pour la mer et pour le littoral, cette stratégie de long terme, doit nous permettre de libérer notre potentiel dans les deux 3 3 domaines majeurs : l'économie, la connaissance, la protection des écosystèmes marins et du littoral, en développant des territoires littoraux et maritime durable est résiliant en soutenant les initiés associative et en levant les freins en promouvant une vision française au sein de l'Union européenne et dans les négociations internationales, cette feuille de route traduit très concrètement on aujourd'hui dans notre territoire, 2 exemples en Bretagne il être là attention que vous portez à la politique maritime national le 1er concerne l'action en faveur du secteur maritime transmanche doublement impactés par le Brexit et la crise du coronavirus en 2020, ce secteur d'activité, a subi un recul de 80 % de son chiffre d'affaires, l'a-t-il Brittany Ferries : la compagnie la plus impactée par ce par cette crise, compte près de 3000 salariés, vous le savez, elle représente un modèle pour notre région, la préservation des emplois et donc une priorité pour le tous les secteurs concernés par ce dossier, j'étais à vos côtés le 18 novembre dernier lorsque vous êtes venu confirmer l'engagement de l'État en faveur de ce fleuron de notre économie, 45 millions d'aides et 16 millions d'euros d'abandon de créances, une aide en partie financé par des fonds européens, il est important de le rappeler, les acteurs économiques du transmanche ont acté le principe selon lequel la crise traversée structurellement bouleverser ce secteur d'activité, une stratégie globale dans le cadre du Fontenoy maritime s'avère donc nécessaire et c'est le sens des travaux que vous menez le second exemple de cette politique maritime qui se concrétise sur nos territoires, porte sur l'intégration du port de Brest Roscoff au saut au réseau central des réseaux transeuropéens de transport en 2013, l'intégration du port à ce réseau était sollicité par les élus et acteurs économiques, le gouvernement nous a entendus et a agi auprès de la Commission européenne pour que ce projet puisse être effectif dès l'année prochaine, c'est une immense victoire pour l'Ouest trop en alliant fret maritime et ferroviaire, ce que le Store maritime préfigure de ce que seront les ports du futur en misant sur la décarbonation, la décarbonation, pardon, des transports, les acteurs politiques et économiques ont unanimement salué ces actions majeures de l'État en faveur de l'aménagement du territoire depuis le 1er janvier la France assure la présidence du Conseil de l'Union européenne le 18 novembre dernier à St Paul de Léon dans le cadre de votre allocation de vos allocution aux Assises de la pêche, vous avez rappelé que cette présidence représentait une occasion unique de faire avancer, voire de finaliser certains dossiers je souhaiterais, Madame la Ministre, attirer votre attention sur 2 dossiers, en particulier le 1er concerne la mise en place des clauses miroir dans nos accords commerciaux, il n'est plus acceptable que les produits alimentaires de la mer importés dans l'Union européenne ne respecte pas les mêmes normes que celles appliquées au sein même de l'Union nos professionnels se heurte depuis trop longtemps à une concurrence déloyale et s'en trouve pénalisée pour vous non, madame la ministre nous dit que nous éclairer sur les ambitions de la présidence française sur ce point particulièrement sensible, le second sujet sur lequel je souhaite attirer votre attention porte sur les attentes des consommateurs et sur le rôle de l'État pour accompagner et être le levier des transitions les consommateurs souhaitent de plus en plus disposer de produits durables répondant à leurs attentes en termes de qualité mais aussi de respect de l'environnement, les acteurs économiques l'ont compris et s'engage, mais il existe encore des freins au développement de certaines filières personne été-moi de nouveau de m'appuyer sur une situation que rencontre notre territoire breton pour illustrer mes propos pour l'importation de produits bio au sein de l'Union, les États membres désignent des postes de contrôles frontaliers à ce jour, seuls 4 ports en France dispose de l'agrément européen qui autorise l'importation de ces marchandises en provenance de pays tiers hors Schengen si l'ensemble des ports bretons est habilité pour l'importation des produits alimentaires non non biologique, aucun d'entre eux ne l'ait à ce jour, référencés pour les produits bio, pourtant de plus en plus d'entreprises locales souhaitent limiter les empreinte carbone la situation actuelle est un véritable non- sens écologique puisque les produits importés par ces entreprises bretonnes parcours jusqu'à 500 kilomètres sur la route, dans ce cadre, le développement d'autorisation permettant d'ouvrir plus de points d'entrée frontalier pour l'importation de marchandises bio dans nos ports français constituerait un signal positif, pouvez-vous, Madame la Ministre, nous éclairer sur la position du gouvernement sur cette question, je conclurai mon intervention sur la tenue à Brest en février prochain du sommet international One Océan, l'objectif sera de définir un cadre réglementaire pour mieux protéger les océans, et en particulier les eaux internationales, des zones de grands fonds très convoité et pour lequel le droit international est quasi inexistant,

je vous remercie et je voulais juste conclure en vous souhaitant à tous et à toutes une très bonne année sur des flots paisible et tranquille. Merci, cher collègue, la parole est à présent Monsieur Pascal Alizart du groupe, les républicains, vous avez ça nous nous chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous évoluons désormais dans un environnement stratégique marqué par l'affirmation de la puissance, le retour du fait accompli et la mise en cause du multilatéralisme et du droit, accélérateur de la globalisation des échanges, la mer redevient un espace de conflictualité où chacun fait valoir ses intérêts les fonds marins représente un terrain de rapport de force avec notamment les câbles sous-marins, la mer, ce sont aussi des Detroit vitaux, entre autres, le Pas-de-Calais, Gibraltar, le Babel montée d'Ormuz Malacca il y en a d'autres, dont il faut continuer à garantir le libre franchissement ainsi la valeur stratégique et économique de la mer s'est accrue en 2017, la revue stratégique relevé que les espaces maritimes sont au coeur des tensions croissantes par leur rôle central dans la mondialisation des flux de toute nature y compris numériques les ressources qu'ils contiennent et le développement des capacités navales et aériennes de frappes à distance le constat, c'est que la Russie par exemple est très présente sur et sous les mers, ces sous-marins viennent régulièrement éprouvé nos moyens et notre détermination sur nos approches maritimes les approches chinoise de production de bâtiments militaires de cartes de navires de commerce et de pêche impressionne et inquiète les routes maritimes de la soie aux objectifs multiples sont une réalité incontournable la Turquie, autre exemple, s'affirme comme une puissance navale en jouant un rôle économique et géopolitique majeur dans un espace qui nous est proche, la Méditerranée après leur pivot asiatique l'empressement des États-Unis à vouloir moderniser et renforcer leur flotte, montre l'importance qu'ils accordent au nouveau grand jeu en mer avec le pacte AUKUS il concourt à la prolifération nucléaire dans le Pacifique, dans ce contexte, les autorités de la marine française souligne régulièrement que ce qui n'est pas protégée et pillé puis contesté et prédisent notamment le retour du combat Naval de haute intensité, l'honneur, mais aussi la difficulté de la France et de disposer d'une façade maritime importante et d'être présente sur toutes les mers du globe, ou presque, car ce sont des territoires, des populations des écosystèmes des richesses naturelles à préserver face à des périls environnementaux des prédateurs désinhibé qui était des contestations de plus en plus forte, en particulier nos territoires ultramarins sont en première ligne face au réchauffement climatique à l'immigration clandestine, au trafic et à la pêche illégale, c'est aussi une concurrence sérieuse en matière d'industrie navale de transport maritime ou de porcs que nous devons affronter lors des débats sur la programmation militaire nous inquiétons des Maliens comtés affectés à la surveillance de nos zones et aux différentes opérations navales les moyens certes ont évolués durant l'exécution de la LPM ne le contexte s'est durcie, pendant ce temps, le monde s'accélère et nous sommes confrontés au défi de la masse, la question du format de la marine, mais aussi de la disponibilité opérationnelle se pose l'avenir du futur avant d'union de patrouille maritime est aussi incertain en océan Indien et dans le Pacifique, nous déployons des bateaux anciens faiblement armés dépourvus d'équipements de guerre électronique et en nombre limité, qui sont en décalage avec les bâtiments récents des Marines partenaires, cela nous renvoie à la stratégie indo-pacifique de la France ambitieux sur le papier, elle se heurte à l'immensité des espaces aux réalités locales et au jeu et au moyen des superpuissances le camouflet subi lors de l'annonce de l'annulation du contrat en Australie et de la conclusion du pacte AUKUS affecté notre crédibilité régionale et internationale, l'entrain mesuré des Européens à nous soutenir, doit nous interroger, quelle sera l'arrêt l'effectivité de la stratégie indo-pacifique de l'Union européenne personne je crois ici ne souhaite que s'inscrivent dans les esprits le principe selon lequel la défense de l'Europe, c'est l'OTAN et la défense de l'indo-Pacifique, c'est la la France mise beaucoup sur le partenariat stratégique avec l'Inde mais l'Inde mise aussi sur la Russie et les membres du quad au 1er rang desquels les États-Unis, comment parler de souveraineté au bout du monde lorsqu'on éprouve les plus grandes difficultés à exercer ses droits face aux voisins britanniques, alors que la présidence française de l'Union européenne, des buts et bientôt le cycle électoral en France, nous sommes face à des défis immenses, il nous faudra les relevés rapidement, sous peine d'un déclassement irréversible et d'un pillage de nos ressources, je vous remercie. Merci, cher collègue, la parole est à présent Madame Hélène Conway Mouret du groupe socialiste, vous avez 4 minutes chers collègues.

Madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous Français, nous entendons par souveraineté la capacité d'agir en toute indépendance sans avoir à nous aligner sur d'autres pays ou d'avoir à obtenir leur aval et faire appliquer le droit français sur tous nos territoires, doté d'un domaine maritime, de plus de 10 millions de kilomètres carré, la France doit surveiller, protéger d'immenses étendues sur tous les océans, celle qui juste nos frontières hexagonales, c'est-à-dire la Méditerranée et l'Atlantique, où se situent les Antilles françaises et la Guyane, mais aussi l'indo-Pacifique où vivent près de 2 millions de Français, le gouvernement a pris dans le cas de la loi de programmation militaire 2019, 2025, des engagements en faveur de la modernisation des capacités de la marine, cet objectif a été en partie atteint, mais notre dispositif aéro-maritime demeure dotée de moyens vieillissant, or au rythme actuel des investissements le renouvellement s'étalera jusqu'à 2030, voire au-delà, pour les frégates de surveillance, il existe une tension constante entre les moyens que nous devons engager pour le maintien de notre souveraineté sur nos espaces maritimes la garantie de la liberté de circulation dans les espaces communs en temps de paix et ce qui serait nécessaire pour la haute intensité dans une action menée en coalition, mais aujourd'hui, nos moyens sont sous tension pour faire face à certaines marines étrangères et leur faible militarisation risque de nous conduire à une incapacité à participer au pot sur défensive mise en place par nos alliés, avec un risque élevé de déclassement militaire le cadre budgétaire à venir sera forcément contraints au vu de l'état de nos finances publiques qu'est-ce qui guidera alors notre choix entre la livraison de torpilles de ravitailleurs de frégates FDI de corvettes, de nouveaux patrouilleurs ou la construction d'un nouveau porte-avions pour faire face à la multiplication des engagements 3 grandes priorités semble émerger. Premièrement, la poursuite des livraisons de nouveaux équipements afin de renforcer nos capacités amphibies intra-Théâtres qui sont actuellement très limité de remplacer nos frégates de surveillance inadapté à l'évolution de la conflictualité et de poursuivent la réalisation du programme abs Simard essentiel pour le contrôle des zones économiques exclusives, il est difficile d'assurer la discrétion d'une flotte en action au vu de la lenteur des déplacements des bâtiments supervision par la 3D Space aérien capteur électronique radar et optiques aéroportée est aussi compliquée par l'étendue des espaces maritimes ces bâtiments de surface sont des proies faciles pour les systèmes à 2 années qui ont été développés en Chine et en Russie, ainsi il serait nécessaire de renouveler la composante de surveillance maritime à la combinant avec un programme de surveillance spatial plus ambitieux, deuxièmement, le respect du droit maritime international à l'heure où celui-ci de plus en plus contesté bafouée et où son socle actuel, la convention de Montego Bay, dont nous fêtons cette année les 40 ans, et de plus en plus remise en cause, l'Europe peut et doit faire entendre sa voix, troisièmement le développement d'une stratégie maritime civil et militaire dans un cadre européen en effet notre domaine maritime nationale donne à lui seul à l'Europe une dimension et une présence mondiale,

et pour la France, 3,5 %. Donc, au vu de l'ampleur de ce réarmement une coopération européenne renforcée s'impose, le programme est européenne Patrol Corvette paraît répondre à la problématique en indo-Pacifique qui nécessite le prépositionnement des bateaux dans cette zone d'où l'importance stratégique de la Nouvelle-Calédonie pour leur mouillage le pacte AUKUS est un autre exemple de la nécessité de se regrouper pour être plus forts menant pourtant 2 premières puissances mondiales pour conclure, s'il est bon d'être ambitieux, écoutons nos militaires qui sont partout en première ligne et agissent de plus en plus au sein de coalitions rendues nécessaires par les moyens engagés face à la montée en puissance technologique et matériels de pays qui ne partagent pas nos valeurs étant à vouloir s'imposer par la force, la réalité est que si nous voulons conserver notre influence, nous devons mettre en adéquation nos ambitions et nos moyens, je fais le voeu qu'à l'avenir, le Parlement soit intimement associé aux futures décisions prises dans le cadre d'une d'un processus mûrement réfléchi pour tout ce qui relève de notre souveraineté et du domaine de la défense, je vous remercie. Merci, cher collègue et ensemble nous finissons ces interventions par notre collègue Didier Mandelli du groupe Les Républicains, vous avez 4 minutes chers collègues. Madame la présidente, madame la Ministre, mes chers collègues, les larmes de nos souverains ont le goût salé de la mer, qu'ils ont ignoré cette citation du cardinal de Richelieu résonne plus que jamais aux oreilles de ceux qui aiment la mer. Avec le développement des échanges, des énergies renouvelables et le potentiel des fonds marins, la mer est devenue l'objet de convoitises et de stratégies de conquête de la part des grandes nations, présent sur l'ensemble des océans, les espaces maritimes sous juridiction française s'étendent sur plus de 10 millions de kilomètres carrés, les orateurs précédents l'ont évidemment évoqué pesant de notre pays, le second domaine maritime le plus vaste du monde derrière les États-Unis cela nous permet de disposer d'avantages économiques et géostratégiques, a priori, malgré cette situation exceptionnelle, notre pays a progressivement tourné le dos à la mer, j'en veux pour preuve l'absence d'un ministre, le ministère de la mer pendant près de 30 ans, la création d'un ministère de plein exercice, c'est une première étape indispensable pour la mise en place et le suivi d'une politique maritime à moyen et long terme, j'appelle de mes voeux à ce que ce ministère message à tous les candidats soient installer définitivement être souverain de son domaine maritime, c'est avoir la capacité de le défendre contre toute forme d'intrusion qui menacerait notre espace où nos infrastructures économiques et militaires, je voudrais évoquer rapidement avec vous quelques sujets très occupation. Dans le cadre du groupe mer et littoral que je préside, nous avons mené une série d'auditions, mettant en lumière de menaces pressantes sur notre souveraineté portuaire nous savons désormais que la Chine, cela a été évoqué également précédemment avec sa stratégie de nouvelles routes de la soie, cherche à développer les interconnexions avec le reste du continent, qu'on appelle eurasiatique, notamment à travers des investissements d'entreprises chinoises dans Les chinoise Cette présence et ça c'est ainsi de plus en plus visible dans les ports européens en Grèce, en Italie, face à cette menace sur l'indépendance de nos infrastructures, aucune proposition ne figure dans la stratégie nationale portuaire, porté par le gouvernement, la protection de notre souveraineté portuaire sera pourtant des enjeux majeurs des années à venir, j'appelle donc de mes voeux, ce qu'un rapport puisse être réalisé sur la réalité de la stratégie chinoise et de son influence sur notre secteur maritime et portuaire, comme le demandait d'ailleurs Michel Vasseur dans sa proposition de loi adoptée au Sénat en décembre 2020. Par ailleurs, nous devons maintenir un regard vigilant sur l'Arctique, symbole des désastres du réchauffement climatique, nous regardons cette partie du monde, peu à peu, disparaître sous nos yeux, tandis que nous observons cette situation d'autres nations comme la Chine, la Russie, les États-Unis réfléchissent déjà à l'exploitation de ces nouvelles routes maritimes, cette situation pose de nombreuses questions et j'appelle à ce que dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, la France puisse porter une véritable stratégie avec les pays riverains afin de garantir la stabilité de la zone, c'était d'ailleurs l'une de vos quatre orientation en 2017 madame la Ministre, enfin la souveraineté économique et militaire doit être également environnemental, bien sûr, nous possédons plus de 57000 kilomètres carrés de récifs coralliens qui font de la France, le second pays dans ce domaine au monde en Nouvelle-Calédonie, où se situe la seconde plus grande barrière récifale au monde en Polynésie ou si tu 20 % des atolls coralliens de la planète, zone de reproduction des espèces et de reconstitution des stocks de pêche, nous avons une responsabilité envers cette biodiversité menacée concernant l'érosion du trait de côte, nous attendons les collectivités locales du littoral attendre de véritables propositions en particulier sur le plan des financements voilà madame la présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues rapidement évoqué les enjeux et défis auxquels notre pays est confronté, il nous appartient de tout mettre en oeuvre ou conforter bien sûr mais surtout renforcer sa place sur cette introduction la souveraineté maritime doit être l'expression de la grandeur de la France, merci de votre attention. Merci, cher collègue, la parole est à présent à Madame Annick Girardin, ministre de la mer.

Madame la présidente, mesdames et messieurs les sénateurs, je vous remercie d'avoir inscrit ce débat à l'ordre du jour. Cela prouve une chose, c'est que la stratégie maritime française reprend la place qu'elle mérite dans les enjeux nationaux j'en suis ravie et ici, dans cette maison, sur les 3 derniers mois, j'ai eu l'occasion, chaque mois, de venir et d'être auditionné sur les questions maritimes cela montre toute l'importance que prend le sujet ici, plusieurs sujets plusieurs questionnements et dans mon intervention dans le temps qui m'est imparti, ce ne sera pas facile de répondre à tous par exemple parler des clauses miroir aussi rapidement que que le temps qui m'est donnée, c'est un peu court et je veux le dire madame la sénatrice Nadège avec nous sommes avec Julien Denormandie, très en accord sur le combat que nous devons mener sur d'cas des accords de libre-échange de lieu sur les clauses miroir, c'est ce que nous continuerons de faire, des informations particulières vous seront données aux uns et aux autres sur les sujets que vous avez ouvert au-delà de l'audition, qui a été la mienne ici le 9 décembre sur le Brexit et la pêche ou le 21 sur les Outre-Mer dans la politique maritime de la France et je serai ici à nouveau le 18 janvier pour être auditionné sur la mission flash sur la protection, l'exploration et l'exploitation des grands enfants, moi, j'ai souhaité vous parlez de la stratégie maritime française que je porte conforter bien sûr notre souveraineté garantir nos intérêts stratégiques et économiques sur les mers et les océans du globe, bien entendu, c'est important et ça s'inscrit pleinement

assure la présidence de l'Union européenne depuis le 1er janvier 22 c'est donc l'occasion de réaffirmer la dimension maritime de l'UE, particulièrement dans un monde qui se durcit, vous l'avez dit les uns et les autres, les arsenaux militaires se développe pour affirmer les les souverainetés avec force les zones de contestation du droit de la mer se multiplient et puis dans le même temps, la lutte contre les activités illicites ou ça n'avait parlé la pêche illégale ou encore la piraterie nécessite une attention constante que les océans sont plus que jamais les supports du commerce mondial, ces menaces à et fragilise la géopolitique des maires la politique maritime du gouvernement forte du retour d'un ministère de la mer de plein exercice, gravitent autour de 3 axes forts notre souveraineté, nos intérêts stratégiques et nos intérêts économiques, nos axes de enfin, les axes de notre politique maritime, c'est d'abord l'affirmation sereine de notre souveraineté, la France reste toujours attaché à l'application pleine et entière de la convention de Montego Bay oui, qui a aujourd'hui 40 ans, madame la sénatrice Hélène Conway Mouret, vous avez raison, il faut le saluer, pour moi la Pierre angulaire du développement pacifique des activités des États en mer, c'est par cette convention, que la France a 31 voisin avec laquelle elle doit s'entendre pour délimiter ses espaces maritimes, j'en profite d'ailleurs pour saluer l'immense travail accompli depuis 10 ans pour moderniser nos décrets de délimitation ils comprennent désormais pour la plupart les coordonnées géographiques précises de nos espaces maritimes que vous pouvez facilement visualiser sur le portail national des limites maritimes qu'on appelle les limites maritimes au pluriel, point gouv point FR, vous pouvez bien entendu consulté en permanence ces données, il nous reste 11 des limitations certains on en parlait, qui ne font pas encore l'objet d'un accord finalisé la France reste toujours ouverte au dialogue avec ses voisins, c'est important, mais dans les cas les plus compliqués, notamment autour de certaines villes françaises et je dis bien certaines îles françaises il y a pour moi aucun doute sur ce point et et je partage vos remarques, monsieur le sénateur Alain Cadec ou encore monsieur Olivier Zico Colautti vous avez raison de dire il faut avoir le courage d'un dialogue franc avec les États, mais qui restent des partenaires pour nous et une autre marque qui pour moi est toujours importante, c'est qu'on dise le mépris n'est donc pas non plus une option pour la France, enfin, pour assurer la surveillance et la maîtrise des activités dans ces espaces maritimes la France déploie sa fonction garde-côtes composée des unités et aéronefs de la marine nationale, des affaires maritimes de la douane des forces de police et bien sûr de gendarmerie ses capacités physiques d'interception voient leurs actions de plus en plus dirigée par le développement des moyens de surveillance satellitaire, je parle des signaux radioélectriques ou encore de l'imagerie radar voire optique, certains d'entre vous m'ont déjà interrogé sur la suffisance de nos moyens pour assurer la surveillance du 2ème espace maritime mondial alors justement ces dernières années, les capacités de la marine nationale ont bénéficié d'une loi que vous connaissez de programmation militaire inédite certains on en parlait après une décroissance qui n'a été stoppée qu'en 2015 le budget de la mission Défense a connu depuis 2017, une remise à niveau sans précédent, passant de 32,3 milliards d'euros à 40,9 milliards d'euros pour 2022, le budget de la marine progresse et vous l'avez rappelé, il y entre 21 et 22 alors je redis avec force ce quinquennat c'est celui qui a fait le plus pour le renouvellement de nos moyens de surveillance en mer, toutes administrations confondues 6 patrouilleurs commandé en Outre-mer 8 commandée pour la métropole et 8, bâtiment d'assistance qui doivent être livrés comme dit vedette côtière des douanes pour la métropole et pour les Outre-Mer, autant de preuves concrètes de notre action, tout cela figure dans le schéma directeur de la fonction garde-côtes au comité interministériel de la mer 2019 par le 1er ministre second axe, celui de notre politique maritime. La garantie de nos intérêts stratégiques dans une approche multilatérale, vous en avez parlé, je l'ai dit, la France reste très attachée aux équilibres de la convention de Montego Bay comme Joël Guerriau je veux réaffirmer ici Monsieur signataires, la liberté de navigation doit rester un principe fort. Par ailleurs, il est de l'intérêt de la France de conserver sa place dans l'industrie câbles hier avec 2 fleurons français a appuyé pour conserver notre souveraineté et exporter notre savoir-faire, je pense bien entendu à Alcatel Submarine Networks ou Orange Orange La haute mer offrent ainsi des droits mais elle impose aussi des devoirs, et j'ai eu l'occasion de rappeler régulièrement nos devoirs c'est pourquoi dans les négociations du traité de la biodiversité en haute mer, ce qu'on appelle Bibi, la France soutient le concept d'océan comme bien commun et nous le redira à Brest en février lors du sommet, un océan voulue par le président de la République, je veux bien entendu ici le redire au sénateur Jacques Fernique, et vous l'avez dit, les connaissances scientifiques sont le préalable incontournable pour déterminer raisonnablement par exemple des aires marines protégées efficace en haute mer. Mais la responsabilité, c'est aussi respecter le rôle de l'autorité internationale des fonds marins. L'AFM pour fixer les règles d'exploration, voire d'exploitation dans la zone des fonds marins sous la haute sous Vous le savez, il y a aussi une question sur la ZES, France 2030, a fait la part belle d'ailleurs ou à la connaissance maritime futur et sachez que j'en suis ravie, nous avons là des grands défis à relever, enfin notre approche, elle est aussi multilatéral de ces questions qui implique de développer des relations de coopération régionale par exemple la France accroît son influence dans l'océan Indien, vous en avez parlé l'axe dos pacifique et bien dans l'océan Indien, en ayant intégré en 2021, à l'unanimité, hein, le Forum des garde-côtes asiatiques et puis plus largement, nous mettons en oeuvre le 14ème Objectifs de développement durable, qui a pour thème de conserver et exploiter de manière durable, les ressources des océans alors ce cet objectif durable numéro 4 heures c'est l'ADN de mon ministère, je l'ai déjà dit et nous le portant portant cette voie également dans les 12 organisations régionales de gestion des pêches dans lesquels nous siégeons, nous la France aux côtés bien entendu aussi de l'Europe, là encore grâce effectivement à nos territoires ultramarins notamment pour atteindre cet objectif, il nous faut d'abord connaître précisément de ressources et il paraît indispensable qu'au XXIe siècle Europe soit en mesure de connaître précisément l'état de ses stocks, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, de tous ses stocks, il nous faut donc une véritable politique de gestion des ressources halieutiques, là encore, c'est un sujet à porter à porter au niveau européen, mais nous avons aussi sur ces sujets à faire mieux, côté français, c'est la des grands objectifs d'ailleurs du plan d'action pour une pêche durable que j'ai proposé au président de la République et qui a été validée le 17 décembre dernier à l'Élysée devant les professionnels de la filière pêche ce plan sera finalisé d'ici la fin du quinquennat et concernera l'ensemble des façades maritimes, y compris bien entendu l'Outre-Mer, je m'y suis engagé ce matin avec l'ensemble des organisations professionnelles, j'ai également l'intention de porter ce sujet à l'occasion de la PFUE bien entendu, pour partager cette vision avec nos partenaires européens et puis pour parler rapidement du dernier axe, celui qui concerne nos intérêts dans l'économie bleue et pour vous dire que la compétitivité du pavillon en France avec la dynamique du Fontenoy du maritime lancée avec les armateurs, il y a maintenant un an, porte déjà ses fruits cette compétitivité elle repose, et vous le savez, sur une stratégie de flotte pour faciliter son financement et la rendent plus écologique, avec le déploiement du suramortissement Vert ou encore la possibilité de coupler le recours au crédit bail avec la garantie interne ou encore la garantie de projets stratégiques selon effectivement sur le positionnement du projet et bien entendu également une action résolue sur l'emploi, l'objectif est bien d'améliorer le parcours et la carrière des marins français, avec la création d'une aide à l'emploi maritime pour 3 ans et avec le doublement du nombre d'officiers qui sortent de formation de l'ANSM d'ici quelques années, enfin, second levier du développement économique et dernier la consolidation des atouts stratégiques constituent nos ports dans toutes leurs dimensions, j'ai entendu Martine ou encore Didier Mandelli en parler et insisté sur cette stratégie portuaire, hé bien, je le redis ici. J'ai un objectif de faire de la France le 1er port européen, bien entendu, dans toutes ses dimensions et, pour cela, il faut d'abord parler collectif et d'avoir cette stratégie globale qui qu'une que nous devons encore affiner je n'oublie pas la croisière qui traverse une période très difficile à cause du Covid les enjeux de l'Hexagone et de ceux d'Outre-mer en pleinement, a été pris en compte dans la stratégie nationale portuaire, la reconquête de parts de marché sur les ports concurrents étrangers se fera uniquement par un développement industriel et logique logistique durable, vous l'avez dit, et j'entend renforcer l'leur l'leur complémentarité, je parle de collectif dans la logique de façade pour conclure, il me reste 3 mots, je voudrais rappeler qu'en mer, il n'existe pas de frontières, mais bien des limites à l'intérieur desquelles l'État côtier développe ses activités dans le respect des libertés des autres en mer l'immobilisme n'est pas permis et je pense vous avoir aujourd'hui assuré ou rassurer sur la détermination de l'action du gouvernement en faveur de sa souveraineté maritime au regard des enjeux stratégiques et économiques, je vous remercie. Merci madame la ministre, mes chers collègues, je vais lever la séance prochaine séance demain mercredi 5 janvier à 15 heures pour les questions d'actualité au gouvernement, la séance est levée, bonne nuit. Merci